Chacun le sait, si notre mix électrique est l'un des moins carbonés du monde, c'est grâce à l'atome. Or, depuis cinq ans, nous ne savons plus où nous en sommes. La baisse de la part du nucléaire à 50 % du mix électrique n'a certes pas été remise en cause, mais l'objectif a été retardé de dix ans. Fessenheim a été fermée, et l'arrêt de quatorze autres réacteurs est encore au programme. Le grand carnage suit son cours, et le plan d'investissement France 2030 va allouer un milliard d'euros au développement des petits réacteurs et des réacteurs de quatrième génération, alors que cet axe de recherche avait été abandonné en 2019 avec le prototype Astrid. Et l'on ne sait toujours pas ce que vous voulez faire de la technologie de l'EPR Monsieur le Premier ministre, en matière de nucléaire, le « en même temps » ne peut plus durer. Très bien ! Sauver les accords de Paris impose de relancer le nucléaire tout de suite, car, sans lui, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif d'une réduction de 55 % des émissions en 2030. À court terme, nous ne pourrons pas décarboner dans les proportions requises sans la pleine puissance des réacteurs actuels, car les SMR () et les éventuels futurs EPR ne seront pas disponibles avant quinze flou, monsieur le Premier ministre ? Comment peut-on afficher de grandes ambitions climatiques et perdre tant de temps sur le nucléaire ? Allez-vous enfin abandonner le projet de fermer des réacteurs pour nous permettre de respecter notre engagement de 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050 ? Quand allez-vous sortir du bois concernant la construction de l'EPR ? La parole

Cette réduction passe d'abord par une baisse de notre consommation énergétique en général : la stratégie nationale bas-carbone prévoit cette diminution de la consommation à hauteur de 40 d'ici à 2030. Elle passe aussi par plus de production électrique, parce que notre électricité est une électricité très largement décarbonée. Elle l'est d'ailleurs parce que, comme la France s'y était engagée, nous avons fermé trois de nos quatre centrales à charbon. La quatrième restera pour sa part en fonctionnement limité tant que l'approvisionnement breton ne sera pas pas assuré par ailleurs. En ce qui concerne le mix énergétique, les scenarii proposés par RTE nous montrent deux constantes : la première, c'est le besoin de continuer à produire de l'électricité, parce que notre consommation d'électricité va augmenter ; la deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables.

Différents scenarii nous montrent aussi l'importance de la place du nucléaire dans ce mix décarboné. C'est la raison pour laquelle la programmation pluriannuelle de l'énergie avait fixé, pour 2035, un horizon de 50 % de nucléaire

le professeur Delfraissy annonce que 20 % des lits des hôpitaux sont fermés faute de personnel, quelle est la réponse du Gouvernement ? « Il faut recompter Toujours le même déni de réalité, le même refus d'écouter médecins, personnels, élus et usagers ! Vous les avez méprisés quand ils tiraient la sonnette d'alarme et que vous poursuiviez vos réductions budgétaires : 17 milliards d'euros ont été économisés sur la santé Vous refusez d'entendre que le Ségur n'est pas suffisant pour répondre au profond malaise actuel. Il est insuffisant sur la revalorisation salariale, insuffisant pour conjurer la dégradation des conditions de travail et de soin Qu'allez-vous faire pour y remédier ? Allez-vous enfin décréter un moratoire sur les fermetures de lits ?

Je ne peux, chère madame, vous laisser dire des choses à ce point inexactes. Vous avez tout à fait raison : la situation de l'hôpital public et de notre service de santé est difficile. Catastrophique ! Mais il vient de faire face, de façon exemplaire, à une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent depuis un siècle. Les personnels de santé sont fatigués,

intervention sont parfaitement exacts. Mais entendons-nous bien, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s'agit pas de fermetures de lits pour cause budgétaire. Les budgets sont là, les postes sont ouverts, mais ils ne sont pas pourvus

Quant au Ségur de la santé, madame la ministre, vous le savez très bien, il représente, pour les personnels comme pour l'investissement, un effort inédit. Il s'agit certes, pour partie,

Quand M. Véran approuvait des budgets de restriction à l'hôpital, j'étais déjà de celles qui se dressaient contre ces politiques, et le groupe CRCE plus encore.

Madame la ministre, en janvier 2021, nous avons débattu dans cet hémicycle de la possibilité d'étendre le RSA (revenu de solidarité active) aux moins de 25 ans. J'avais défendu l'idée selon laquelle l'accompagnement vers l'emploi et l'émancipation était l'outil le plus efficace pour répondre aux besoins de notre jeunesse. Ma position demeure inchangée. Je me félicite donc que le Président de la République ait annoncé hier matin la création d'un nouveau dispositif d'aide pour les 500 000 jeunes les plus éloignés de l'emploi. Dans la lignée du plan « 1 jeune, 1 solution » et de la garantie jeunes dont il s'inspire, un contrat d'engagement permettra d'accompagner vers l'emploi des jeunes sans travail ni formation, qui souvent se trouvent en situation de très grande précarité. Beaucoup a été fait ces derniers mois. Trois millions de jeunes ont trouvé un emploi, un parcours d'insertion ou une formation grâce au plan « 1 jeune, 1 solution » depuis son lancement. Le niveau d'embauche des jeunes s'est quant à lui maintenu, malgré la crise, grâce aux primes à l'embauche et à l'alternance. Pourtant, trop de jeunes demeurent sur le bord de la route. En France, près de 20 % des jeunes sont aujourd'hui au chômage. Dans certains départements d'outre-mer, ce taux avoisine les 50 %. C'est évidemment beaucoup trop. Le dispositif que vous proposez, madame la ministre, est ambitieux. Pouvez-vous nous en préciser les contours et les objectifs ? Qu'apportera-t-il de plus que la garantie jeunes, dont le nombre de bénéficiaires n'a cessé d'augmenter ces dernières années ? Comment s'opérera la bascule entre ces deux dispositifs ? Enfin, quels moyens financiers et humains seront mobilisés en 2022, et dans les années qui suivent, pour assurer l'efficacité de ce programme ?

comme vous l'avez souligné, avec le développement inédit de l'apprentissage, l'investissement dans les compétences et, plus récemment, le plan « 1 jeune, 1 solution », la jeunesse est le fil rouge de notre action depuis 2017. Tout va bien ... Toutes ces politiques portent leurs fruits. Malgré la crise sanitaire, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi est au plus bas depuis 2008. Pourtant, certains jeunes risquent de ne pas profiter de la reprise et de rester durablement éloignés de l'emploi. Nous nous démarquons du reste de l'Europe par un taux de jeunes ni en emploi, ni en formation, ni en études qui reste trop élevé, particulièrement dans certains territoires d'outre-mer, comme vous l'avez rappelé. C'est pour cela que nous mettrons en oeuvre, dès le 1 mars 2022, le contrat d'engagement jeune, destiné aux 500 000 jeunes durablement éloignés de l'emploi. Nous leur proposerons un accompagnement personnalisé et intensif entre 15 et 20 heures par semaine, assorti d'une allocation pour ceux qui en ont besoin. Le contrat d'engagement jeune a vocation à remplacer la garantie jeunes en capitalisant sur l'expérience des missions locales. Nous voulons également tirer parti de toutes les solutions du plan « 1 jeune, 1 solution », qui viendront enrichir les parcours. Je pense par exemple aux immersions en entreprise pour découvrir un métier, aux formations qualifiantes dans les secteurs en tension ou aux remises à niveau sur les compétences de base. En deux mots, monsieur le sénateur, le contrat d'engagement, c'est du gagnant-gagnant. Pour les jeunes, c'est la possibilité d'accéder à l'autonomie grâce à un emploi. Pour les entreprises, c'est la possibilité de trouver le salarié ou l'apprenti dont elles ont besoin. Ce n'est

l'observation des conditions de vie (Crédoc) en octobre, les périodes de confinements et de restrictions d'activité ont conduit quatre millions de nos compatriotes à basculer, sinon dans la grande pauvreté, du moins dans une situation très préoccupante de fragilité. Ces « nouveaux vulnérables » ont un profond sentiment de déclassement ils travaillent dur et doivent reporter, ou à y renoncer, des dépenses essentielles de santé, d'équipement, d'alimentation, voire de logement. Dans le même temps, l'écart salarial entre les femmes et les hommes continue de se creuser cette année, celles-ci occupent 80 % des emplois à temps partiel et en sont les premières victimes. Tous les jours, les associations d'aide aux plus démunis nous alertent sur l'explosion des demandes alimentaires, surtout chez les jeunes. Quant à la baisse du chômage, elle cache une réalité cynique : elle s'est faite au prix d'une flexibilité du droit du travail et d'une précarisation des emplois, venant gonfler ainsi le nombre de travailleurs pauvres, faute d'une rémunération, d'une stabilité ou d'un temps de travail suffisants. Madame la ministre du travail, comment peut-on accepter aujourd'hui, en France, que les gens qui travaillent dur ne s'en sortent pas ?

Monsieur le sénateur Pla, bien évidemment, nous n'acceptons pas que certains travailleurs puissent ne pas vivre dignement de leur travail. C'est notamment pour cela que, depuis des mois, dans le cadre de l'agenda social que nous avons lancé avec le Premier ministre au mois de juillet 2020, nous avons mis au coeur de nos discussions la situation des travailleurs de la deuxième ligne, tous ces travailleurs qui avaient été mis en lumière par la crise, qui connaissent trop souvent des conditions de travail et des conditions d'emploi que leur rémunération ne permet pas de compenser. Je pense effectivement aux secteurs de la propreté ou de la sécurité. permettre aux négociations de s'engager dans les branches, j'ai chargé deux expertes de faire la lumière sur les conditions de travail et de rémunération dans ces secteurs. invité les organisations patronales et syndicales à lancer des discussions visant à améliorer la situation de ces travailleurs de la deuxième ligne, dont, je le redis, nous avons pu voir toute l'utilité dans la crise.

le bas niveau de rémunération de nombreux salariés de ce pays tient non pas au taux horaire du SMIC, mais à la fragmentation à l'extrême des contrats de travail, à la précarisation des contrats de travail. C'est bien contre cette précarité du travail que nous voulons lutter grâce à la réforme de l'assurance chômage. C'est raté

Vous avez beau tordre les chiffres dans tous les sens, madame la ministre, vous n'arriverez pas nous faire croire que ce sont les ménages les plus modestes, notamment les précaires, qui ont été les grands bénéficiaires de votre réforme, de toutes les réformes d'ailleurs. Car, depuis la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ce qui progresse, c'est l'épargne des riches et la précarité chez les plus pauvres. Vous savez, pour amuser le peuple,

! Croyez-moi, les travailleurs n'attendent pas des étrennes électorales ni des négociations de branche ; ils veulent des résultats et des solutions durables, de suite. La réalité, madame la ministre, c'est que les travailleurs pauvres d'aujourd'hui sont condamnés à devenir les retraités pauvres de demain

agricole, impulsée par le groupe RDSE, et dont j'ai été la rapporteure aux côtés du président Jean-Marc Boyer conclusions, après de nombreux déplacements sur le terrain et de nombreuses auditions. Un trait caractéristique résume nos impressions : le dynamisme. Le dynamisme des apprenants, avec lesquels nous avons échangé : ils sont porteurs d'envie et d'espoir pour notre agriculture, mais aussi plus largement pour la vitalité des territoires ruraux. Le dynamisme des personnels, qui ont toujours à coeur d'innover et de délivrer un enseignement d'excellence, comme le démontrent les résultats obtenus lors des examens, les meilleurs de toutes les filières. Le dynamisme des responsables des différentes fédérations d'enseignement, qui s'efforcent d'adapter constamment

Au terme de ce travail, nous sommes plus que jamais convaincus que l'enseignement agricole, qui doit impérativement rester dans votre giron, monsieur le ministre, est l'outil indispensable pour nos filières agricole et alimentaire, pour nos jeunes, pour nos terroirs, en métropole comme dans les outre-mer. Pourtant, cet outil remarquable est aujourd'hui fragilisé, par les contraintes budgétaires, par l'agribashing, parce qu'il n'est pas assez valorisé par le système d'orientation et qu'il souffre d'une réelle concurrence avec l'éducation nationale, parce que nos agriculteurs n'ont pas encore une juste rémunération. Nous estimons que l'enseignement agricole a besoin de perspectives nouvelles, d'un véritable projet stratégique et de moyens à la hauteur des enjeux. Vous avez annoncé certaines réformes, nous le reconnaissons, mais nous souhaitons que vous alliez plus loin. Saisissez-vous des 45 propositions de notre rapport pour offrir des perspectives de long terme à l'enseignement agricole ! Nos jeunes le méritent, l'avenir de notre agriculture en dépend. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part aujourd'hui de vos intentions ? La

Nathalie Delattre, permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre rapport, à la fois pour sa qualité et pour son contenu. Je remercie également le président Boyer et l'ensemble de vos collègues- je les

Ainsi, les émissions accidentelles de méthane tout au long de la filière d'exploitation et de distribution du gaz naturel fossile fragilisent fortement le bilan carbone du gaz par rapport au charbon. ne permettent pas d'en faire, en aucune manière, une réponse efficace à la crise climatique. Certaines villes américaines, par exemple, engagées sur le climat, refusent aujourd'hui de développer des réseaux de gaz. Or,

En clair, « on intègre vos centrales à gaz dans la taxonomie des investissements verts au niveau européen »- ce qui ouvre l'accès quand même au financement de 200 milliards d'euros du pacte Vert pour l'Europe -, en échange de quoi « vous nous aidez à y intégrer aussi du nucléaire français Ce deal se ferait clairement sur le dos du climat. En conséquence, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous démentir clairement, simplement et catégoriquement l'existence, l'idée même, d'un tel pacte contre-nature ?

repose sur le charbon. Il est absolument nécessaire, vital même, de sortir de ce charbon, qui est vraiment très

que ces installations ne devraient fonctionner que de manière temporaire. On estime à moins de 22 % du temps sur une année ce recours en cas de pointe. Je vous confirme que le gouvernement français a toujours défendu le fait que le nucléaire avait sa place parmi les énergies décarbonées. De fait, avec 50 % de notre mix électrique assuré par le nucléaire à horizon 2035,

franchement, s'il fallait ouvrir toutes grandes les vannes du gaz fossile russe pour trouver les milliards de la relance du programme nucléaire français, vous auriez quand même bien du mal à faire avaler ensuite l'histoire- la fable - d'un nucléaire français allié du climat La parole est à M. Joël Guerriau, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. nous sommes le 3 novembre. Il y a très exactement un mois, le 3 octobre 2021, le gouvernement algérien annonçait qu'il interdisait désormais à l'aviation militaire française de survoler son territoire. territoire. Ces vols étant à destination du Sahel, vous comprenez à quel point ils sont importants dans le cadre de notre lutte contre le terrorisme. Il se trouve que nous avons 5 000 soldats qui, au quotidien, interviennent pour lutter contre le terrorisme au Sahel.

cette suspension n'a pas d'effets directs sur nos opérations. Les avions de chasse, les avions de transport tactique, les drones qui opèrent au Sahel décollent tous, pour l'essentiel, du Niger. En ce qui concerne les vols militaires qui décollent depuis le territoire national pour rejoindre l'opération Barkhane, je vous confirme qu'ils survolent, en général, le territoire algérien. Il s'agit majoritairement de vols de relève militaire et il se trouve que nous sommes en mesure, lorsque cela est nécessaire- et c'est nécessaire en ce moment -, d'emprunter d'autres routes aériennes. Vous l'avez souligné vous-même, monsieur le sénateur, ces itinéraires de contournement ont nécessairement un coût. Ils ont un coût humain, ils ont un coût matériel, ils ont un coût en carburant. Ce coût, nous le suivons évidemment avec la plus grande attention.

je ne sous-estime pas, évidemment, la portée symbolique de cette décision et, j'insiste devant vous, je la regrette. L'Algérie est en effet un voisin de notre espace méditerranéen, c'est aussi un partenaire crucial dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ; sa connaissance approfondie de la région, ainsi que des dynamiques locales, est particulièrement précieuse. j'espère que cette situation prendra fin rapidement et que nous pourrons reprendre un dialogue plus apaisé sur ces enjeux de sécurité majeurs pour nos deux pays. La parole

interdits de passage au-dessus de l'Algérie, est complètement incohérent et inacceptable. J'espère, madame la ministre, que vous arriverez à convaincre nos interlocuteurs algériens de revenir sur cette décision. J'aimerais honnêtement que l'on sache très exactement quel est son coût, car je pense que ce dernier s'élève à plusieurs millions d'euros,

J'ai lu, comme certains d'entre nous, madame la ministre, le livre de Daniel Rosenweg sur les organismes de complémentaire santé, communément appelés mutuelles. L'auteur en dénonce les « dérives, les défaillances et les dysfonctionnements ». En dix ans, les tarifs de ces organismes ont augmenté de 45 %. Actuellement, près de 11 millions de nos concitoyens doivent avoir recours à l'aide de l'État pour s'offrir une complémentaire santé. C'est devenu un produit de luxe. Pire, en 2020 et 2021, alors que la pandémie a réduit les dépenses de santé des mutuelles

qui bénéficient de contrats négociés, et, de l'autre, les retraités et les indépendants, qui payent très cher des contrats individuels tout en étant moins bien couverts. Une fois encore, les frais de gestion sont pointés du doigt. À 21 %, ils représentent quand même 8 milliards d'euros. Ils atteignent 40 % dans certains contrats. Ainsi, sur 1 000 euros cotisés, 400 partent en frais administratifs. Est-ce normal d'investir dans des courses de voile, dans des concerts, des vignobles, des marathons et autres publicités télévisuelles ? Que comptez-vous faire, madame la ministre, pour assainir cette situation, intolérable quand il s'agit de santé ?

que les prestations qu'elles prennent en charge. Nous sommes soucieux des tarifs payés par les plus fragiles, notamment les seniors. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduits à mettre en oeuvre des réformes telles que la complémentaire santé solidaire ou le « 100 % santé », qui ont des impacts concrets sur le coût des soins assumé par nos concitoyens. Dans notre pays, chaque personne peut désormais bénéficier d'une solution dentaire, auditive ou visuelle adaptée, sans frais plus personne n'a à choisir entre bien voir ou bien entendre. C'est un progrès social majeur, une avancée décisive, notamment pour nos concitoyens les plus modestes. Pour autant, dans ce contexte, nous pouvons aussi nous interroger sur l'impact des frais de gestion des mutuelles, qui évoluent à la hausse quand ceux de l'assurance maladie sont en baisse, ou en tout cas stables. La crise a d'ailleurs révélé que seule une intervention publique permettrait la prise en charge rapide à 100 %, en tiers payant, des dépistages de la vaccination et des téléconsultations. Ces constats doivent nous interroger sur l'articulation la plus efficiente entre assurance maladie obligatoire et complémentaire. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie expertise, en ce moment même, différents scénarios d'évolution, dont l'un d'entre eux consiste à créer une grande « Sécu », qui couvrirait de manière simple et lisible, intégralement d'ailleurs, le panier de soins. Il s'agit là de travaux qui n'engagent

Comme l'a rappelé l'éminent président Longeot, la France s'est fixé, voilà cinq ans, lors des accords de Paris, des objectifs ambitieux. Mais rappelez-vous aussi qu'en début d'année, ici même, nous avons eu un débat sur un risque de blackout énergétique. fermé Fessenheim et acheté en Allemagne de l'énergie produite dans les conditions que l'on sait. Absolument ! Qu'en est-il cette année ? Comment comptez-vous tenir les objectifs

sur cette situation, que le Gouvernement suit évidemment, en lien avec RTE, le réseau de transport d'électricité, et les principaux opérateurs des outils de production. Au printemps 2021, RTE a présenté ses analyses en matière de sécurité d'approvisionnement pour les prochains hivers dans son bilan prévisionnel à l'horizon 2030,

La sécurité d'approvisionnement progresse toutefois légèrement chaque hiver jusqu'en 2024, avec la mise en service de nouveaux moyens de production. Je pense à l'EPR de Flamanville, mais aussi aux renouvelables, notamment les parcs éoliens en mer., cette sécurité d'approvisionnement s'améliorera significativement, au point que les marges deviennent positives par rapport aux critères de risque de défaillance à l'horizon 2025. Pour cet hiver spécifiquement, les analyses de RTE seront complétées par une mise à jour, qui sera vraisemblablement publiée dans la seconde moitié de novembre, ce qui nous permettra un point à date. Pour l'hiver prochain, EDF continue d'optimiser son programme de maintenance pour maximiser la disponibilité du parc nucléaire, notamment avec une évolution du nombre de tranches nucléaires disponibles en janvier et février, ce qui améliorera notre visibilité. Par la gestion prudente de l'ensemble des moyens de production, en particulier des réservoirs hydrauliques, nous permet également de maximiser la capacité de production disponible, l'état de remplissage des barrages étant très satisfaisant. l'appel d'offres effacement pour l'année 2022 a été lancé par RTE fin juillet, après approbation du cahier des charges par le ministère de la transition écologique. Il nous autorise à disposer de capacités de flexibilité supplémentaires à partir de janvier 2022. Nous sommes donc tout à fait vigilants, mais très confiants sur ces différents critères. J'ai écouté avec attention la lecture de vos fiches, madame la secrétaire d'État. Chacun sait vos tergiversations sur le nucléaire. Pour notre part, nous sommes au clair sur la question. Alors que c'est un atout pour notre pays, vous avez le nucléaire honteux, aigri. À vouloir se passer du nucléaire, on va finir par éteindre toutes les lumières. Vous voulez 100 % de véhicules électriques, mais vous voulez vous passer de la principale source d'électricité, et ce n'est pas votre trop-plein d'éoliennes qui suffira. La France des campagnes leur dit non La France des campagnes, comme la France des villes, peine à se chauffer. La France des campagnes peine à rouler pour travailler, alors que c'est sa seule solution de mobilité. Pour sortir de l'impasse, « l'énergie pour tous » passe par une baisse massive des taxes L'État y gagnera à court terme,

Le président Emmanuel Macron, fidèle à sa stratégie d'autosatisfaction, y a vanté son action tout en mettant en cause les pays retardataires. Cette posture de donneur de leçons passe mal, car la France, sous votre gouvernance, vient d'être condamnée pour carence fautive dans la lutte contre le changement climatique. Sous votre gouvernance, nous avons été le seul pays européen du G20 à augmenter nos financements fossiles depuis l'accord de Paris. Sous votre gouvernance, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été respectés, et vous avez refusé, dans la loi Climat, pourtant texte phare de votre quinquennat, de vous aligner sur le niveau de réduction de l'Union européenne. Président de la République a même relevé les plafonds d'émission autorisés ! Sous votre gouvernance, en coulisses des négociations sur le projet européen de classification des énergies, la France manoeuvre pour faire reconnaître le gaz comme une énergie verte. Votre gouvernement promet de consacrer 6 milliards d'euros par an aux pays du Sud, mais la plupart de ces fonds seront encore accordés sous forme de prêts, et non de subventions, creusant davantage leur dette. En résumé, votre gouvernement tient des doubles discours tout le temps et partout ! Après le climato-scepticisme, voici le climato-cynisme Alors, monsieur le ministre, à quand une cohérence entre vos paroles et vos actes ? À quand des mesures fortes et un budget vert pour un véritable tournant écologique ? La

J'y serai moi-même demain, et, vous l'avez rappelé, le Président de la République s'y est rendu lundi, pour l'ouverture de la COP26. Madame la sénatrice, sous notre gouvernance,

sur lequel nous n'étions que très peu nombreux à nous mobiliser au niveau européen au début du quinquennat, a finalement été largement partagé par tous les pays européens. Aujourd'hui, c'est la norme c'est la norme européenne et c'est elle qui donne le signal de la mobilisation pour la bonne réussite de la COP26. Blabla. Sous notre gouvernance, nous sommes passés de zéro milliard d'accompagnement aux pays en développement dans l'accord de Paris à 7 milliards d'euros, contribuant ainsi à une mobilisation qui a permis, sur l'initiative du Président de la République, à Rome, le week-end dernier, d'atteindre les 100 milliards d'euros en faveur de la lutte pour l'atténuation et l'adaptation. Sous notre gouvernance, nous avons fait passer une loi, que vous n'avez pas votée, qui permet d'agir pour la résilience et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je regrette au passage que vous ne l'ayez pas votée. Sous notre gouvernance a été voté un plan de relance, qui permet de mobiliser 30 milliards d'euros pour la transition écologique. Sous notre gouvernance, un plan d'investissements un plan d'investissements d'avenir a été annoncé par le Président de la République, permettant de nous donner les moyens d'accomplir les engagements que nous prenons

Monsieur le ministre, nous ne sommes pas étonnés de votre réponse. Évidemment, vous avez tout bien fait et votre action est irréprochable. Cependant, vous avez été condamnés pour inaction climatique. Personne n'est dupe, la France n'est pas à la hauteur

Comment diffuser cela quand tant de femmes dans le monde, et même en Europe, sont menacées ou persécutées dès qu'elles tentent de se découvrir ? Quelle grave dérive, monsieur le ministre ! L'islamisme n'avance pas seulement par la terreur. En Europe comme en France, il cherche à s'installer dans les institutions chargées de défendre la liberté. Et il y parvient Doit-on y voir la marque de la Turquie d'Erdogan, toujours membre du Conseil de l'Europe, ou des organisations islamistes, comme les Frères musulmans, qui tentent depuis des années d'imposer des programmes de recherche et d'agir sur nos institutions ? Comment accepter ce détournement des fonds publics des démocraties pour normaliser non pas une liberté religieuse, mais un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté, un interdit d'égalité, un interdit de fraternité ? L'Europe, si prompte à remettre en question les valeurs de certains États membres, ne peut pas être le cheval de Troie de l'islam politique. Alors, monsieur le ministre, envisagez-vous des sanctions ? Comptez-vous agir en cessant, par exemple, de siéger temporairement au Conseil de l'Europe et de participer à son financement ?

Je note que cette campagne choquante pose un double problème. D'une part, un problème procédural, puisque les visuels publiés sur les réseaux sociaux société civile lors d'un atelier consacré spécifiquement aux discours de haine à l'encontre des personnes de confession musulmane. Le fait qu'ils aient été relayés par le compte twitter du service antidiscrimination du Conseil de l'Europe entretient l'ambiguïté

passés et par les réactions qu'elle a suscitées, a, de fait, conduit au résultat inverse de celui qui était recherché, et a gravement méconnu les principes sur lesquels est fondée notre approche du sujet. C'est pourquoi, madame la sénatrice, nous avons, dès hier, fait part de notre désapprobation- les tweets ont été retirés -et nous avons aujourd'hui demandé à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe de confirmer publiquement la suppression de ces messages.

vous vous opposez systématiquement à nos propositions pour la France. Je pense à l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, les mineurs, ou encore au burkini. Je croyais que votre quinquennat était placé sous le signe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pourtant, je constate un renoncement supplémentaire et une incohérence. Je regrette que nous n'envoyions pas un bon message aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi la parole de la France est respectée, puisque cette campagne continue toujours. La

Au début de l'été, la Russie a pris une décision qui contrevient aux intérêts de notre pays, en obligeant les producteurs de champagne à apposer la mention « vin pétillant » sur leurs bouteilles et en n'autorisant la mention « champanskoïé », soit champagne en russe, que sur les vins effervescents fabriqués en Russie. Récemment, nous avons obtenu un sursis de quelques semaines, jusqu'au 31 décembre. C'est trop court ! L'appellation champagne, protégée dans 120 pays, répond à des critères très précis d'élaboration et de production qualitatives dans une zone géographique répartie sur cinq départements la Marne, l'Aube, l'Aisne, la Haute-Marne et la Seine-et-Marne. Rappelons qu'en 2015 la communauté internationale a reconnu le caractère unique et exceptionnel de la Champagne, en l'ajoutant à la liste de l'Unesco. La Russie, fière de son histoire, doit reconnaître la singularité de notre histoire champenoise. Les appellations d'origine contrôlée et protégée européennes apportent des garanties d'authenticité aux consommateurs européens comme russes. La France respectera les appellations du tvorog ou de la smetana russes. Aussi, La Russie doit respecter ses engagements internationaux et reconnaître qu'« il n'est champagne que de la Champagne

le Gouvernement est mobilisé pour défendre les exportateurs, tout comme les indications géographiques et les appellations protégées. Quand nous avons appris que la Russie avait adopté une loi qui privait nos producteurs de la faculté de recourir au mot champagne en alphabet cyrillique sur les étiquettes à l'arrière des bouteilles de champagne, tout en leur permettant de maintenir la dénomination champagne sur les étiquettes principales à l'avant des bouteilles, nous nous sommes tout de suite mobilisés. Nous avons, avec Julien Denormandie, rencontré les producteurs pour calibrer notre réaction et coordonner notre action. Nous nous sommes d'ailleurs rendus dans la Marne, votre département, À la demande du Premier ministre, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Julien Denormandie et moi-même avons saisi nos homologues russes pour leur faire part de nos préoccupations. Notre action a porté ses fruits, puisque, le 26 octobre dernier, les autorités russes ont pris la décision d'appliquer un moratoire sur cette loi jusqu'au 31 décembre

Monsieur le ministre, votre présence à Épernay, accompagné de M. Denormandie, a sans nul doute compté pour obtenir ce moratoire, mais c'est insuffisant. Vous l'avez bien compris. Le 31 décembre, c'est demain ! N'oublions pas qu'une telle mesure peut concerner prochainement toutes nos appellations.

Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, depuis plusieurs mois, nous vivons la libération de la parole sur les violences sexuelles, notamment celles qui sont faites aux enfants. Régulièrement, nous sommes confrontés à l'horreur ; une prise de conscience salutaire se réalise dans notre société. Je tiens à saluer ici les travaux importants réalisés au Sénat par la mission commune d'information présidée par Catherine Deroche sur la pédocriminalité. La semaine dernière, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a rendu un premier avis, sur les mères en lutte. mères en lutte. Cet avis est éclairant : il met en avant toute la problématique qui s'impose aux parents dès lors qu'un enfant fait le choix de libérer sa parole. C'est pourquoi la Ciivise a formulé trois recommandations fortes pour mieux protéger les enfants. Nous le savons aujourd'hui, la parole des enfants n'est que trop peu écoutée et entendue. Nous savons également que très peu d'enfants s'expriment et que la réalité des faits est bien au-delà des plaintes que l'on connaît. Chaque année, 22 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles. Or, en 2020, moins de 2 000 personnes ont été poursuivies pour viol ou agression sexuelle à caractère incestueux. Trop fréquemment encore, en 2021, le syndrome d'aliénation parentale est mis en avant, notamment lors des dépôts de plainte. toutes les études soulignent l'inexistence factuelle d'une telle dynamique. Ce concept conduit pourtant trop souvent les professionnels à ne pas prendre en compte le témoignage des enfants et les risques de violences auxquels ils sont exposés. L'Espagne s'est déjà engagée contre le recours au concept d'aliénation parentale et le Parlement européen a récemment fait part de sa préoccupation sur le sujet. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, sur la base de ces recommandations, que compte faire le gouvernement français ?

les travaux de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, que j'ai installée dès le 1 août 2020- et non en janvier dernier à la suite de la publication du livre de Camille Kouchner -, parce que la lutte contre les violences, notamment sexuelles, faites aux enfants est une action prioritaire de ce

mères en lutte. Le troisième objectif de la Ciivise était enfin de formuler des recommandations de politique publique pour que nous, décideurs- et je sais à quel point le Sénat travaille sur ces questions -, puissions améliorer la protection des enfants dans notre société.

le sénateur, le syndrome d'aliénation parentale. Dès 2018, le garde des sceaux avait émis une circulaire à l'attention des magistrats pour leur préciser que ce syndrome n'était ni reconnu ni justifié. Vous parlez aussi de libération de la parole des enfants on le sait, la qualité du recueil de la parole est, elle aussi, cruciale dans ces affaires, notamment pour éviter les classements sans suite. C'est la raison pour laquelle, d'ici à l'année prochaine, nous créerons 100 unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Pour conclure, je profite de votre question, monsieur le sénateur, pour vous annoncer que, conformément à la demande du Président de la République du 23 janvier dernier,

je vous remercie, mais je pense que ce gouvernement doit arrêter le « en même temps » et rapidement passer des paroles aux actes ! Rendre la justice quand un enfant révèle les violences qu'il a subies est certes une mission délicate, mais c'est un devoir moral collectif, qui n'est pas contraire au principe fondamental de la présomption d'innocence.

Ce contrat s'adresse seulement à 400 000 jeunes sans emploi ni formation ; il met donc de côté 600 000 d'entre eux, auxquels s'ajoutent les étudiants qui connaissent de grandes difficultés. Il exclut aussi les jeunes qui enchaînent les contrats courts sous-payés et tourne ainsi le dos à cette jeunesse précaire qui a la volonté de s'en sortir, mais qui subit la crise. En trois mois, l'enveloppe a fondu ; le nombre de bénéficiaires, quant à lui, a été divisé par deux et même par dix ; c'est la révélation du jour ! En effet, si l'on exclut les jeunes déjà pris en charge par les dispositifs existants, seuls 100 000 nouveaux entrants seraient en fait concernés. Les logiques budgétaires ont repris le dessus ! Alors, madame la ministre, outre l'effet d'annonce, quel sera le nombre réel de nouveaux entrants ? Pouvez-vous nous confirmer que les dispositifs actuels comme la garantie jeunes et l'accompagnement renforcé, qui accueillent 300 000 jeunes, n'ont pas vocation à être pérennisés, mais qu'ils vont se fondre dans le nouveau dispositif, ce qui impliquerait la création de seulement 100 000 nouvelles places ? Enfin, quels moyens en formation et en accompagnement

je ne suis pas sûre, voyez-vous, que l'on progresse beaucoup au service de l'insertion professionnelle des jeunes en s'envoyant des chiffres à la figure ! Ce que je peux vous dire, monsieur le sénateur, c'est qu'il y a 1 million de jeunes dans notre pays qui ne sont ni en emploi ni en formation. Pas plus que vous je ne m'en satisfais.

Ces réponses, à l'évidence, capitalisent sur ce que nous faisons depuis plus d'un an, avec notamment le plan « 1 jeune, 1 solution », dont je rappelle qu'il a permis à plus de 3 millions de jeunes de trouver un emploi, une formation,

retour à l'emploi. Nous voulons aussi multiplier la possibilité pour les jeunes de trouver une réponse sur le territoire. Il convient donc que ce contrat soit proposé non seulement par les missions locales, mais aussi par Pôle emploi et par les associations de lutte contre la pauvreté, avec lesquelles nous travaillons. Les moyens seront là : nous venons de déposer un amendement

je comprends votre malaise : il y a eu des effets d'annonce, mais en 24 heures on a divisé le nombre de bénéficiaires par deux ! La jeunesse de France est un investissement d'avenir. Elle a besoin qu'on lui fasse confiance et qu'on ne la suspecte pas de se complaire dans un assistanat.

qui est pour les Anglais un sujet éminemment symbolique, puisqu'il s'agit de souveraineté maritime. Je rappelle que l'accord sur la pêche a été obtenu aux forceps et au prix de certaines concessions, 24 heures avant un tant redouté. À cette heure, je considère néanmoins que le gouvernement français a fait preuve de naïveté en imaginant que nos ex- partenaires au sein de l'Union européenne allaient respecter l'accord signé. Aujourd'hui, les Britanniques refusent, en violation de l'accord, de délivrer à la France les licences de pêche dans l'arc Manche-mer du Nord, plus particulièrement autour des îles anglo-normandes et dans le détroit du pas de Calais. Contrairement à leurs affirmations, les informations disponibles concernant les navires éligibles leur ont pourtant été transmises. On voit donc bien que les Britanniques font preuve dans cette affaire d'une extrême mauvaise foi. Madame la ministre, nous n'y comprenons plus rien ! La semaine dernière, Clément Beaune, le poing ferme, nous annonçait un ultimatum et des mesures de rétorsion à l'égard du Royaume-Uni. Or, il y a 48 heures, le Président de la République proclamait une reculade molle Par ailleurs, nous constatons à travers ce dossier que la France se trouve bien isolée, puisque les autres membres de l'Union européenne ne se précipitent pas pour nous soutenir, alors que la présidence française de l'Union européenne commence dans quelques semaines à peine. Alors, madame la ministre, que pouvez-vous nous dire sur cette situation ?

est bien mis en oeuvre. Vous en avez été le grand témoin, tout simplement parce que nous avons régulièrement eu des débats avec l'ensemble des élus des différents territoires concernés. De par votre territoire, de par votre expérience et de par votre connaissance de ces sujets,

très élevés, qui affectent leur compétitivité. Un mécanisme permet de limiter l'impact de ces augmentations. Il s'agit de l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui

Tous les industriels français ne pourront faire valoir leurs droits ; ils devront finalement, après écrêtement imposé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), acheter leur électricité sur le marché de gros à des prix pouvant atteindre 130 euros du kilowattheure,

On a récemment appris qu'EDF, entreprise détenue à plus de 80 % par l'État, avait perdu 400 millions d'euros en spéculant sur les marchés de l'énergie. Pour le consommateur, la facture ne cesse de croître. Pensez-vous, madame la ministre, que l'État, actionnaire majoritaire, a joué son rôle de contrôle ? Allez-vous, à l'avenir, laisser EDF spéculer ainsi ? La

pas sur la situation de ces derniers : le Premier ministre a annoncé des mesures fortes, notamment un chèque inflation de 100 euros, qui concernera 38 millions de Français. Mais nous avons également agi pour les entreprises.

aujourd'hui la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le foncier agricole

l'impact de cette concentration sur la démocratie ». L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

tous ici. Certains amendements visent à modifier un grand nombre d'alinéas, sur des sujets très différents, et sont donc incompatibles avec d'autres amendements, de telle sorte que, sans examen séparé, nous prenons le risque de nous perdre dans de très longues- trop longues -discussions communes. Afin de faciliter le bon déroulement des débats, j'ai proposé ce matin en commission des affaires économiques qu'une demande d'examen séparé de quatre amendements soit formulée en séance. La commission a voté ce matin en faveur de cette demande, sans aucune opposition. En application de l'article 46, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des affaires économiques demande donc l'examen séparé, à l'article 1, de l'amendement n° 19 rectifié de Mme Chantal Deseyne, afin qu'il soit discuté avec l'amendement n° 96, ainsi que des amendements n 177, 59 rectifié

Merci,

Si nous pouvons être fiers du modèle agricole français aujourd'hui, c'est aussi parce que nos aînés ont su développer des outils de politique foncière particulièrement forts et audacieux. En miroir de la politique agricole commune (PAC), cette politique constitue le deuxième pilier du développement agricole qu'Edgard Pisani et ses successeurs ont su construire, en amont d'un troisième pilier que nous sommes en train d'édifier autour de la revue des régimes assurantiels et de couverture des risques climatiques, dont j'aurai l'honneur de discuter avec vous dans cet hémicycle

de l'agriculture, de conserver un modèle agricole de taille humaine, capable de fournir des produits de qualité et de maintenir des hommes et des femmes dans nos territoires, donc permettant le renouvellement des générations.

Le premier enjeu de cette proposition de loi est donc de moderniser et d'adapter nos outils de régulation foncière. Il ne s'agit en aucun cas de s'opposer à la forme sociétaire, mais nous savons tous qu'il y a un trou dans la raquette concernant le contrôle de la transmission des parts sociétaires.

Je sais que nos jeunes agriculteurs et leurs représentants nous regardent attentivement aujourd'hui et je connais les immenses espoirs qu'ils fondent dans le nouveau dispositif que nous allons collégialement créer.

L'absence de régulation des cessions de parts de sociétés agricoles peut en effet limiter notre capacité à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Sur le fondement de ce constat, la proposition de loi consacre un nouveau régime d'autorisation s'appliquant aux opérations de prise de contrôle des sociétés détenant ou exploitant du foncier. Il s'agit d'une procédure spécifiquement adaptée aux contraintes du marché sociétaire, complémentaire du contrôle des structures et de l'action des Safer. Le texte qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, est le produit de riches débats, d'abord à l'Assemblée nationale, puis en commission des affaires économiques au Sénat.

étant, nous devons aujourd'hui adopter des dispositions qui ne vident pas le texte de sa pertinence et ne rendent pas le dispositif inopérant dans les faits. De ce point de vue, permettez-moi de partager avec vous mes inquiétudes au regard de certaines évolutions du texte adoptées en commission au Sénat. Il me semble en particulier indispensable et prioritaire de conserver le caractère opérationnel de la procédure. Nous le devons au monde agricole et je sais que nous ferons collectivement tous les efforts nécessaires pour parvenir à un texte précis et calibré sur ce point. Les Safer doivent rester, en tant qu'elles proposent des analyses et des solutions de compensation, au centre du dispositif. J'assume pleinement cette volonté. Elles sont depuis soixante ans les structures consacrées à la dévolution du foncier sous toutes ses formes. J'ai noté que vous aviez beaucoup échangé sur le rôle des Safer lors de l'examen du texte en commission. Le choix qui a été fait de confier l'instruction des dossiers aux Safer est celui de la simplicité et de l'efficacité. Je pense que la proposition

Nous le verrons lors de l'examen de vos amendements, plusieurs acteurs alertent sur le rôle jugé trop prépondérant des Safer dans la nouvelle procédure. Je partage votre souhait de veiller à ce que notre niveau d'exigence envers elles soit à la hauteur des responsabilités que le législateur pourrait leur confier-

nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le foncier agricole se situe au carrefour de plusieurs politiques publiques la terre, monsieur le ministre, mes chers collègues, est la raison d'être et l'outil de travail de nos exploitants agricoles est le support de l'installation de jeunes agriculteurs ; elle est surtout une véritable ressource naturelle, socle de biodiversité et garante de notre souveraineté alimentaire. n'a pas attendu 2021 pour se pencher sur le foncier agricole, mais, comme pour tout pan de la législation, il nous revient, à nous, parlementaires, de prendre à échéances régulières un peu de recul sur le modèle français et d'examiner ce qui fonctionne et ce qui doit être complété ou renforcé pour nous adapter aux temps que nous vivons. Le recours croissant à des sociétés dans le secteur agricole est l'une de ces évolutions récentes qui appellent à réviser notre droit. C'est pourquoi cette proposition de loi est la bienvenue.

S'il y a urgence, monsieur le ministre, qu'attend donc le Gouvernement pour nous présenter, comme s'y était engagé le Président de la République voilà cinq ans, une loi foncière ambitieuse et cohérente ?

Nous sommes ici face à une double spécificité française. La première tient au grand nombre de sociétés agricoles. Environ 36 % de nos exploitations sont constituées sous forme sociétaire, contre 5 % en moyenne dans les autres États de l'Union européenne. Les transactions sociétaires sont aussi et surtout les plus significatives : elles représentent environ 7 % des transactions et près de 20 % de la valeur du marché foncier agricole. Quant aux échanges de lots, ils concernent des surfaces et 90 hectares, environ dix fois supérieures à celles qui sont échangées directement entre personnes physiques. La seconde spécificité tient à l'impératif de renouvellement des générations. Alors que près d'un tiers de nos agriculteurs partiront à la retraite dans les dix prochaines années, l'accès au foncier agricole demeure l'un des principaux freins à l'installation d'agriculteurs. L'enjeu est de taille, mais la situation actuelle empêche d'y répondre de manière satisfaisante. d'abord, les outils de régulation existants ne permettent d'appréhender que partiellement et de façon imparfaite les transactions sociétaires sur le marché foncier agricole. de contourner les dispositifs de contrôle en vigueur. Ensuite, si des mécanismes de régulation visant à lutter contre l'accaparement des terres agricoles ont déjà été proposés, ils ont régulièrement été censurés par le Conseil constitutionnel, soit parce qu'il s'agissait de cavaliers législatifs soit parce qu'ils portaient atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété. J'ai tenu compte, dans mes travaux, de cet historique législatif. L'équilibre entre libertés constitutionnelles et régulation du marché foncier n'est pas toujours facile à trouver.

Dans cette nouvelle procédure de contrôle, le préfet devrait autoriser individuellement chaque transaction sociétaire susceptible de conduire à une concentration excessive. Cette proposition structurante dépasse de loin la seule rustine d'urgence

Dans ce contexte, j'ai souhaité aborder l'examen de cette proposition de loi dans un esprit de mesure, d'équilibre et de concertation avec mes collègues. que je défends, s'il ne modifie pas les grandes lignes du dispositif de contrôle initialement proposé, apporte tout de même les garanties, les garde-fous et les ajustements nécessaires pour le rendre plus légitime, plus opérationnel et plus acceptable. Premièrement, j'ai souhaité recentrer le dispositif sur l'objectif annoncé de lutte contre l'accaparement et la concentration excessive Le dispositif proposé n'a pas vocation à contrôler toutes les transactions sociétaires sur le marché foncier agricole. Il est en effet indispensable de préserver une certaine fluidité sur ce marché. Économiquement, la concentration n'est pas toujours une mauvaise chose, et le recours à des formes sociétaires présente certains avantages. En revanche, ce qui n'est pas souhaitable, c'est la constitution d'exploitations agricoles de taille disproportionnée, ou encore la spéculation foncière. C'est dans pareils cas que nous pouvons parler d'accaparement des terres et de concentration excessive. C'est cela, et seulement cela, qui doit être combattu par le biais de cette proposition de loi. Dans cette perspective, j'ai notamment souhaité relever le seuil plancher de l'agrandissement significatif, car des exploitations agricoles dont la surface correspond à la moyenne régionale ne sauraient être regardées comme excessives. J'ai également insisté sur la nécessité de préserver la fluidité des transactions qui interviennent dans un cadre conjugal et familial, car nous partageons toutes et tous la volonté de permettre à nos exploitations familiales de se transmettre et de se maintenir. Il m'a également semblé important d'assouplir le dispositif prévu pour les reprises d'exploitation par des associés, actionnaires ou salariés qui travaillent depuis plusieurs années au développement de l'entreprise. Deuxièmement, j'ai souhaité territorialiser davantage le dispositif de contrôle pour rapprocher la décision administrative des territoires et des agriculteurs, en privilégiant une décision du préfet de département plutôt que du préfet de région. Si le seuil d'agrandissement demeure fixé par le préfet de région, j'ai souhaité maintenir la possibilité pour ce dernier de fixer ce seuil à un échelon infrarégional. Troisièmement, j'ai été guidé par le souci d'éviter de placer les acteurs dans des situations délicates, voire risquées. En effet, je suis convaincu de la nécessité de prévoir des garde-fous supplémentaires afin de protéger les Safer d'éventuels conflits d'intérêts, d'asseoir la légitimité de leur intervention et de garantir la transparence de la procédure,

le rôle des Safer dans l'instruction des dossiers me semble finalement incontournable. Tous les auditionnés s'accordent à dire, en effet, que les services préfectoraux n'ont plus les moyens d'instruire seuls et que les Safer disposent d'une expertise essentielle.

Dans cette perspective d'encadrement, la commission des affaires économiques a supprimé la possibilité pour les Safer d'intervenir commercialement et directement sur les dossiers qu'elles auront instruits. Il s'agit selon moi du principal problème du dispositif initial : une même entité ne saurait être à la fois instructrice d'une demande d'autorisation, intéressée financièrement à la mise en oeuvre d'opérations commerciales sur ces mêmes dossiers, et exemptée elle-même de tout contrôle. De manière complémentaire, j'ai souhaité encadrer davantage les mesures compensatoires qui peuvent être demandées par le préfet à des sociétés en contrepartie de l'obtention de l'autorisation administrative. Il ne s'agit en aucun cas d'un affaiblissement du dispositif, mais plutôt d'une mesure de bon sens. J'insiste sur ce point, car il est essentiel : toutes ces mesures adoptées en commission des affaires économiques visent à renforcer le dispositif en clarifiant les rôles de chacun des acteurs concernés. Enfin, j'ai souhaité ajouter l'obligation d'une évaluation complète et précise à trois ans du dispositif de contrôle proposé. Les résultats de cette étude tiendront lieu de clause de revoyure, permettant d'opérer d'éventuels ajustements pourquoi pas, nous l'espérons, dans le cadre d'une grande loi foncière. Voilà donc les positions que je défends au nom de notre commission ; elles se résument en quatre points : recentrer, territorialiser, encadrer et évaluer. La parole

la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires n'a malheureusement pas réussi à pallier la défection du Gouvernement : celui-ci n'aura jamais proposé de grande loi foncière agricole au cours des cinq dernières années, et ce en dépit de la recommandation de la Cour des comptes, des préconisations de la mission d'information commune de l'Assemblée nationale sur le foncier agricole et du caractère essentiel de ce sujet pour la préservation de notre modèle d'agriculture. Nos terres agricoles représentent en effet une ressource particulière, soumise à des tensions et à des convoitises multiples : artificialisation, concentration excessive des exploitations et accaparement par des capitaux aujourd'hui essentiellement français, mais déjà un peu étrangers et risquant de le devenir majoritairement demain. Or, bien que notre pays ait été pionnier en matière de régulation de l'accès au foncier agricole, la création d'outils comme les Safer et le contrôle des structures, il existe une différence de traitement entre, d'un côté, les exploitants agricoles installés à titre individuel et, de l'autre, le format sociétaire, parfois utilisé pour échapper à toutes les contraintes. Cette inégalité s'avère problématique, puisque le contrôle des structures porte exclusivement sur le droit d'exploiter et non sur la prise de participation financière dans une société. S'agissant de contrôler les cessions de titres sociaux portant sur des sociétés et d'agir pour l'installation et la consolidation des exploitations existantes, la présente proposition de loi partait d'une bonne intention. auteurs optent pour un parti pris qui ne peut nous convenir : au lieu de créer un système identique s'appliquant à tous les agriculteurs et à toutes les structures sans distinction, on construit un système parallèle au système actuel, propre au régime sociétaire.

Je reviendrai sur trois points en particulier qui nous posent question : le seuil surfacique de déclenchement du contrôle prévu par l'article 1 ; la latitude laissée aux Safer, extrêmement contraintes dans le texte de la commission ; la question du contrôle des opérations familiales qui, sans remettre en cause l'agriculture familiale, doit faire l'objet d'une vigilance relative si l'on veut éviter la concentration excessive des terres agricoles. Face à la volonté délibérée de la commission d'assouplir le texte pour le libéraliser davantage grâce à une augmentation significative du seuil d'agrandissement et à une multiplication des dérogations au dispositif de contrôle, nous avons donc défendu les propositions suivantes. Dès l'article 1, le seuil surfacique de déclenchement du contrôle a cristallisé les débats. Pour mémoire, la taille moyenne des surfaces exploitées est passée de 28 hectares en 1988 à 62 hectares en 2016, entendu que les exploitations sociétaires utilisent en moyenne trois fois plus de surface qu'une exploitation individuelle. Nous pensons donc que l'objectif général du nouveau chapitre consacré au contrôle des sociétés dans le code rural et de la pêche maritime doit s'apprécier dès le premier hectare. Pour lutter contre le risque de dérives et de détournements offert par les multiples dérogations, nous proposons un seuil de contrôle commun, donc un dispositif équitable et simple, ce qui est souhaité par une grande partie de la profession.

dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), ce qui nous paraît totalement déconnecté de l'objectif de lutte contre la concentration excessive des terres.

Faute d'une véritable définition de ce que l'on entend par actif agricole - et il faudra bien un jour, monsieur le ministre, apporter une réponse à cette question -, participer à la vie de l'exploitation nous paraît la moindre des choses pour bénéficier de l'exemption, et cela doit redevenir une obligation Encore n'évoquerons-nous pas ici le travail délégué et toutes les conséquences délétères qu'il engendre, pour ce qui est en particulier du renouvellement générationnel et du risque d'une agriculture sans agriculteurs. Je voudrais rappeler quelques chiffres éloquents, qui donnent un aperçu du chemin inquiétant que prend notre agriculture : entre 2010 et 2016, le nombre d'exploitations agricoles individuelles a diminué de 19 %, quand celui des exploitations sociétaires n'a cessé de croître, tout comme l'agrandissement des exploitations. Or ce texte, tel qu'il est issu des travaux de la commission, représente un pas supplémentaire vers le capitalisme agricole et la libéralisation à outrance de notre agriculture, à l'opposé des attentes d'une majorité de notre population, laquelle aspire aujourd'hui à une agriculture à taille humaine, respectueuse des sols et pourvoyeuse de productions saines.

Nous souhaitons, à ce propos, rétablir la dérogation, supprimée en commission des affaires économiques du Sénat, bénéficiant aux sociétés foncières agricoles d'utilité sociale. Nos propositions, qui tendaient vers davantage d'équité, d'équilibre et de contrôle réfléchi, n'ont pourtant pas, pour l'instant, été entendues par la majorité sénatoriale de droite. Et du centre ! Nous espérons que les débats à venir- ils seront, je n'en doute pas, riches, passionnés, et probablement longs - corrigeront en partie ces égarements.

Depuis 2017 - notre ministre peut en témoigner -, nous nous attaquons aux causes profondes des dysfonctionnements du modèle agricole. Cela prend du temps et exige des ajustements, mais, au bout du compte, notre modèle est en train de se renforcer. Je fais ainsi référence aux États généraux de l'alimentation et aux deux lois qui en sont issues, visant à refonder totalement les négociations commerciales au profit de nos agriculteurs. Mais penser à l'agriculture, c'est penser aussi à anticiper et à susciter de nouvelles vocations, car le constat est alarmant un agriculteur européen sur deux a aujourd'hui plus de 55 ans, et partira donc à la retraite ces prochains mois. Le renouvellement des générations est par conséquent un impératif. impératif. Le foncier agricole doit donc être plus accessible. La lutte contre l'artificialisation des sols est un premier combat à mener et, à cet égard, une série de mesures ont été votées lors de l'examen du projet de loi Climat Mais ce qui nous réunit cet après-midi, c'est la volonté d'agir contre la concentration des terres. Et il y a urgence ! Le nombre d'exploitations ne cesse de baisser. Quelques chiffres assez parlants peuvent l'attester : en 1955, il y avait 2,3 millions d'exploitations agricoles ; en 2016, il n'en restait que 440 000. C'est le résultat d'une politique agricole de cogestion, de concentration, d'industrialisation des terres et de nos produits. Cette politique a donné des résultats, mais elle n'est plus adaptée à la nécessité d'une agriculture pragmatique, protectrice et ambitieuse.

L'auteur de la proposition de loi s'est donc entretenu, des mois durant, avec les organisations interprofessionnelles, afin d'aboutir à un dispositif qui puisse satisfaire l'ensemble des parties. L'idée est de donner aux Safer les outils qui leur permettront de contrôler les cessions de parts de sociétés et d'agir pour favoriser l'installation de nouveaux exploitants. Ainsi, toute cession au profit d'un acquéreur détenant des terres agricoles au-delà d'un certain seuil sera contrôlée. Ce sera ensuite aux préfets d'autoriser ou non la transaction. Mais notre commission des affaires économiques a considéré, dans sa majorité, que les pouvoirs des Safer étaient excessivement étendus. De fait, une série d'amendements adoptés la semaine dernière ont visé à amoindrir leurs compétences - je fais référence aux mesures compensatoires. note, ici où là, des dérives, celles-ci restent maîtrisées et sanctionnées. Je rappelle que les Safer sont des opérateurs utiles pour nos agriculteurs, qu'elles ne seront jamais décisionnaires et que seul le préfet autorisera ou refusera la cession de parts. C'est en ce sens que nous déposerons des amendements de rétablissement, et nous espérons que la majorité sénatoriale comprendra notre message. Globalement, nous nous entendons tous pour agir : nous souhaitons tous attirer les jeunes générations autour de l'objectif consistant à reconstruire un maillage d'activités et de liens sociaux qui redonne vie à nos territoires. Nous tenons donc à ce que les projets fonciers agricoles à dimension biologique ou écologique puissent être facilités- tel sera l'objet d'un autre amendement de rétablissement présenté par notre groupe, visant les projets à haute valeur sociétale, sociale et écologique. Mes chers collègues, certes, nous le voyons, des divergences de points de vue se font jour, notamment sur les manières d'aboutir, mais nous partageons tous une même ambition : faciliter l'acquisition de nos terres agricoles. Dès lors, continuons à travailler ensemble et trouvons des portes de sortie dans l'intérêt de notre agriculture

en février 2020, notre groupe avait organisé dans ce même hémicycle un débat intitulé : « Foncier agricole : les outils de régulations sont-ils toujours pertinents ? » Nous avions conclu notre débat sur la nécessité absolue d'apporter des ajustements législatifs à notre système régulant le foncier agricole. Le texte proposé par notre collègue député Jean-Bernard Sempastous, dont je salue le travail, tend à répondre à l'urgence de la situation. Urgence, en effet, car de nombreux départs en retraite vont intervenir dans les prochaines années : près d'un agriculteur sur deux fera valoir ses droits à la retraite Nous avons la chance, dans notre pays, d'avoir des jeunes motivés, désireux de s'installer. Il faut donc les aider et faciliter la transmission à leur profit. encore, car il faut surmonter les difficultés actuelles pour accéder au foncier, qui est pourtant le support indispensable de tous les projets agricoles. Les outils de régulation existants ont été mis en place dans les années 1960. Force est de constater qu'ils ne sont plus adaptés pour faire face aux nouvelles manières d'accéder au foncier. Une grande loi foncière est attendue, et même annoncée, depuis des années. Beaucoup l'appellent de leurs voeux. Il faut néanmoins admettre que nous n'en avons pas tous la même définition.

Le champ de ce texte est certes très circonscrit ; il a toutefois le mérite de cibler les pans qui sont aujourd'hui les moins bien régulés. En effet, actuellement, seule l'acquisition directe de terres agricoles par des exploitants ou des sociétés

afin d'atteindre des tailles porteuses d'avenir et de compétitivité économique, mais aussi faciliter la transmission et le renouvellement des générations. La commission a instauré la territorialisation du contrôle en confiant au préfet de département la décision d'autoriser ou de refuser une prise de participation sociétaire ; on rapproche ainsi la décision des territoires. Au regard de la diversité des exploitations, l'échelon départemental sera parfaitement adapté. Par ailleurs, le texte renforce le rôle des Safer en leur octroyant davantage de missions.

En mettant en place un système de contrôle flexible et adapté aux réalités de terrain, ce texte contribue à faciliter l'accès au foncier, que ce soit en propriété ou en location, et à encourager le renouvellement des générations, concourant ainsi à garantir notre souveraineté alimentaire. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que d'autres sujets non présents dans ce texte, d'une importance

pour le renouvellement des générations, donc pour le développement d'une agriculture à taille humaine, pourvoyeuse de valeur ajoutée et d'emplois. Il y a là un enjeu essentiel pour la vitalité de nos territoires pour la sécurisation d'une alimentation locale diversifiée et de qualité. Un accès partagé à la terre est aussi un levier de promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement puisque, bien souvent, on observe une corrélation entre la taille d'exploitation et la qualité de la biodiversité. Si la régulation du foncier agricole doit permettre la nécessaire transition agroécologique, de failles législatives et l'arrivée de fonds spéculatifs dans le secteur agricole se traduisent par des accaparements de terres néfastes pour notre agriculture et pour notre société.

foncière qui était promise par le Gouvernement. Nous aurions souhaité aborder le travail à façon, source de concentration de terres. De même, l'accaparement par des investisseurs étrangers des montages sociétaires n'est pas traité. Ensuite, bien que cette proposition de loi soit présentée comme une avancée dans un contexte d'urgence, non seulement elle ne va pas assez loin, mais elle pourrait s'avérer contre-productive, en particulier dans sa rédaction

en légitimant un contrôle plus faible des agrandissements réalisés des parts de sociétés, elle acte un « deux poids, deux mesures » entre personnes morales et personnes physiques. Elle risque ainsi de décrédibiliser toute volonté régulatrice en créant un système peu efficace

pour les biens passés par le régime d'autorisation créé par le texte. Nous nous opposons aussi à la suppression de l'article 5, qui représentait selon nous une véritable avancée permettant de lutter contre les agrandissements excessifs. Nous sommes ici en désaccord profond avec la commission, qui considère la concentration des terres comme bénéfique, car nécessaire à la compétitivité, ainsi qu'il est écrit dans le rapport. Selon nous, la course à l'agrandissement des fermes est synonyme de perte d'emplois, de valeur ajoutée de biodiversité ; elle est source de difficultés pour de nombreux porteurs de projets, dont certains sont contraints de renoncer, faute d'accès au foncier. La terre est est un bien commun, il est important de le rappeler, base de notre système nourricier. C'est pour cette raison que nous souhaitons construire un système transparent et juste permettant une régulation foncière accordée à nos objectifs en matière d'installation et de consolidation des exploitations. On a beaucoup parlé de liberté : c'est ici la liberté d'entreprendre du plus grand nombre que nous souhaitons défendre et, à travers elle, la transition agroécologique. Nous nous opposerons- hélas ! -à ce texte nécessaire, mais largement insuffisant. La parole est à M.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, parce que la terre est la ressource du vivant, la question de la régulation et de l'interventionnisme public dans la gestion du foncier agricole est déterminante. La question foncière est au coeur du renouvellement générationnel en agriculture, alors que 37 % des paysans vont quitter leurs terres dans la décennie qui vient. Elle doit donc être intégrée à la préparation de la relève, par exemple les aides à l'installation des jeunes agriculteurs. La question foncière est aussi au coeur des problématiques environnementales et de préservation de la qualité des sols et de l'eau. Elle est au coeur d'un modèle d'agriculture de taille humaine, de proximité, que nous souhaitons préserver et développer. Ce n'est pas un hasard si ce sujet complexe a fait l'objet de nombreux rapports ces dernières années et devient peu à peu une préoccupation citoyenne. Au-delà de la question de l'artificialisation, c'est aujourd'hui la concentration foncière qui est en jeu du fait de la fragilisation des outils de contrôle de la propriété et de l'usage des espaces agricoles. En effet, la question foncière n'est plus essentiellement l'affaire des agriculteurs ; elle devient celle d'investisseurs capitalistes et de spéculateurs financiers dont les stratégies de maîtrise du foncier agricole sont totalement étrangères aux objectifs de la politique foncière mise en place au milieu du XX siècle.

Cette proposition de loi soulève donc une question essentielle : comment répondre à l'essor d'une agriculture de firmes et d'une financiarisation des terres qui se font au détriment du modèle agricole ? ? L'accaparement des terres agricoles entraîne en effet la concentration d'une ressource essentielle dans les mains de quelques-uns, au détriment des paysans privés de terre, des jeunes agriculteurs, mais aussi de l'ensemble de nos concitoyens, tant cette question a partie liée avec l'exigence d'une alimentation saine et de qualité. Mon sentiment malgré tout, nous pouvons nous accorder sur deux points. Aujourd'hui, la législation foncière est opaque et incapable de maîtriser la marchandisation de la terre. En outre, l'usage partagé de cette ressource ne peut pas être régulé par les seules lois du marché. Mais la solution proposée ne nous convainc pas. Loin de renforcer les outils de régulation existants, le texte instaure un nouveau régime de contrôle du phénomène sociétaire qui risque de fragiliser encore davantage les formes de contrôle existantes, voire d'accélérer un mouvement de financiarisation qu'il faudrait au contraire combattre. La proposition de loi a un champ trop limité, le déclenchement du contrôle étant doublement conditionné : il faut que la cession de parts conduise à la prise de contrôle d'une société à hauteur de 40 % des droits de vote et que la surface totale détenue après l'acquisition de la société dépasse un seuil d'agrandissement significatif fixé par le préfet de région. Or ces deux seuils, ainsi que les différentes exemptions prévues par le texte, limiteront fortement les opérations soumises au contrôle. Pis, le texte permet de dépasser le seuil d'agrandissement en contrepartie de mesures compensatoires. Dès lors, on peut se demander si cette nouvelle procédure de contrôle n'aura pas un effet contraire à celui qui est recherché, certains se servant de ce nouvel outil pour constituer des sociétés qui permettront de contourner le contrôle des structures. Nous regrettons enfin qu'en lieu et place d'une grande loi foncière nous débattions d'une proposition de loi enserrée dans le temps de l'initiative parlementaire. L'accumulation de petites réformes nuit à la cohérence et à la clarté et témoigne d'un manque de vision globale concernant une thématique pourtant fondamentale. En ce sens, ce texte est une occasion manquée. Il ne répondra malheureusement pas aux objectifs de relocalisation alimentaire, de protection de l'environnement, de défense des droits à la terre et à l'installation. La terre n'est pas un bien comme les autres et il faudra beaucoup plus d'ambition pour la préserver et l'arracher au phénomène de financiarisation, qui nuit à la souveraineté alimentaire et à la biodiversité. Très bien

Malgré notre déception de ne pas avoir à légiférer sur la grande loi promise, nous sommes nombreux à soutenir l'ambition des auteurs de ce texte. Ainsi, mercredi 20 octobre, la commission des affaires économiques approuvé la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Nous en avons d'abord accepté les grandes lignes, car elle répond au besoin de régulation du foncier agricole, qui, rappelons-le, est rongé depuis des décennies au profit de zones commerciales, de lotissements ou d'aménagements de transport. Ses auteurs tentent par ailleurs de répondre à d'autres objectifs, que l'on retrouve notamment à l'article 1 favoriser l'installation des jeunes, lutter contre les concentrations excessives et encadrer l'accaparement des terres. S'y exprime le souhait de maintenir le modèle agricole français, qui est majoritairement de type familial, des chefs d'exploitation dirigeant tout en participant à leur mise en valeur. Aujourd'hui, de plus en plus de terres sont acquises et transmises par le biais de sociétés. Toutefois, les opérations réalisées échappent en grande partie à la régulation. Ce texte s'avérait donc nécessaire.

Lorsque cette proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale, le 26 mai dernier, elle nous était annoncée comme parfaite, ne nécessitant aucun aménagement, car elle ferait l'unanimité. C'est dans cet état d'esprit que nous avions entamé nos travaux voilà quelques mois. Mais le Sénat, après avoir confronté ses analyses à la réalité des auditions de terrain menées dans nos différents départements, a vite compris que l'unanimité autorevendiquée était friable et que des évolutions devaient intervenir. Défendant une posture « de mesure et d'équilibre », notre assemblée a calibré ce texte afin de le recentrer sur ses objectifs et d'y apporter les garde-fous nécessaires : en assurant la territorialisation de la procédure de contrôle, pour rapprocher la décision du terrain et la faire redescendre au niveau du préfet de département ; en relevant le seuil de surface considérée comme excessive afin de focaliser le dispositif sur les objectifs annoncés de lutte contre l'accaparement foncier et la concentration excessive prévoyant une évaluation qualitative et quantitative du dispositif sous trois ans, afin, le cas échéant, de faire évoluer la procédure et d'organiser une remontée d'informations précieuses sur les dynamiques du marché foncier agricole

Sans ambiguïté, elles se sont voulues rassurantes. Placés sous le contrôle du conseil d'administration et des commissaires du Gouvernement, les comités techniques constituent la cheville ouvrière de l'action foncière menée par les Safer pour apporter au plus près des territoires la réponse la plus adaptée aux enjeux identifiés localement et couvrir l'ensemble des missions de service public.

d'une grande loi foncière à l'occasion d'un débat demandé par le groupe Les Indépendants. Cette déclaration faisait écho au projet de loi foncière annoncé en 2019 par le Président de la République, lors de l'ouverture du salon international de l'agriculture. Dans cette grande loi, nous aurions abordé l'artificialisation des sols, le statut du fermage, la transmission des exploitations familiales, la fiscalité associée, etc.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel regret ! Oui, comme mes collègues l'ont dit précédemment, quel regret que la loi de réforme foncière annoncée n'ait pas vu le jour.

d'exemple, dans mon département de l'Hérault, en trente ans, 25 % de la surface agricole utile ont été sacrifiés sur l'autel de l'urbanisation. Quand on sait que certaines terres avaient bénéficié de fonds publics pour l'irrigation, quel gâchis !

En matière de foncier agricole, c'est toute une démarche qu'il convient de repenser. Plusieurs textes ont déjà été adoptés pour tenter d'améliorer le dispositif. Souvenons-nous : en 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt crée un nouveau droit de préemption des Safer.

France, 64 % des exploitations seulement sont individuelles, contre 95 % en Europe. La commission des affaires économiques a proposé de confier aux préfets de département l'instruction des dossiers. Cette territorialisation colle à la réalité du terrain.

préconisait en effet le renforcement de la représentation des collectivités territoriales dans les conseils d'administration des Safer et un encadrement plus strict des pouvoirs coercitifs dont elles disposent. Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur la question du seuil de déclenchement du dispositif de contrôle, qui devrait faire débat au regard du nombre d'amendements déposés sur le sujet

Il faudrait également redonner plus de fluidité à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation. Cela passe par le retour à une consultation seulement facultative des organisations professionnelles, ou encore par la possibilité d'auditionner les parties à la seule appréciation des comités techniques des Safer.

plus de transactions foncières agricoles effectuées par des sociétés échappent au contrôle des Safer ou le contournent. Ainsi, entre 2016 et 2019, 9 % des sociétés ayant cédé des parts ont vu leur capital intégralement transféré des cessions partielles échelonnées dans le temps, sans possibilité pour la Safer d'exercer son droit de préemption,

terres. Cette pression foncière et financière entraîne une difficulté particulière pour les agriculteurs, notamment ceux qui veulent s'installer et n'héritent pas d'une exploitation ou encore ceux dont l'équilibre économique est fragile : celle d'avoir à supporter la charge de l'acquisition du foncier. La structuration familiale des exploitations françaises évolue avec la progression des sociétés agricoles, ce qui conduit à déconnecter propriété foncière et exploitation. La tendance est à la concentration des terres au profit de structures dont tout ou partie du capital peut être financé par des personnes ne participant pas au travail agricole, le risque d'une financiarisation s'en trouvant accru. La question du partage et de la gestion des utilités foncières relance le débat relatif à l'utilisation du territoire français, patrimoine commun de la Nation, et au rôle stratégique que jouent les espaces agricoles là où il s'agit de garantir notre souveraineté alimentaire et de lutter contre l'effet de serre,

que l'instruction de la demande d'autorisation par les Safer, qui conforte leurs missions dans la transparence, et le rôle confié au préfet de département, seule autorité administrative à délivrer l'autorisation, ce texte

Pour reprendre une métaphore chère au général de Gaulle, « si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. » En agriculture, fleuron de notre économie,

Le temps du débat parlementaire est déjà fortement contraint- l'examen en quatrième vitesse de cette proposition de loi en est, ce soir, une nouvelle illustration. C'est pourquoi nous ne saurions aborder sereinement ce débat sans nous exprimer pour présenter la réforme que nous aurions voulu voir mener au travers de cette proposition de loi.

Comme nous l'avons dit en discussion générale, nous sommes très dubitatifs sur les effets réels de cette proposition de loi en matière de lutte contre l'accaparement des terres et contre la concentration excessive,

nous estimons que ce nouveau système pourrait même desservir l'objectif initial du texte, en incitant à créer des sociétés pour bénéficier d'un contrôle plus souple et plus perméable.

Ce dispositif similaire pour tous, soutenu par le groupe socialiste du Sénat comme par celui de l'Assemblée nationale, aurait été le véritable gage d'équité et de simplification que nos agriculteurs ne cessent de réclamer.

Il ne saurait y avoir deux poids, deux mesures, sinon à institutionnaliser une injustice manifeste et à encourager les moins vertueux à choisir le mécanisme le plus opportun pour mieux contourner le système. Le second, l'amendement n° 79, visait à abaisser le seuil de déclenchement du contrôle tel que l'article 1 proposé prévoyait une définition de ce qu'il faut entendre par « prise de contrôle », à savoir « la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale [ ...] le contrôle de la société La proposition de loi initiale fixait ce seuil à 25 % des droits de vote ; afin de tenir compte d'un risque d'inconstitutionnalité relevé par le Conseil d'État, il a été augmenté à hauteur de 40 %. Si nous avons bien pris connaissance des inquiétudes du Conseil d'État, nous considérons néanmoins que ce seuil de 40 % est trop élevé et qu'un contrôle devrait être exercé dès 25 %.

restructurer des exploitations en limite de zones urbaines ; faire respecter le cahier des charges par les acheteurs ou investisseurs qui bénéficient de prix et de droits préférentiels en fonction du bail restant ; faire

de refus. Il s'agit d'un amendement de cohérence : c'est bien le préfet de région qui est l'autorité compétente pour délivrer des autorisations d'exploiter. Aussi convient-il de s'interroger sur la compétence du préfet de département

au motif que ces organismes sont déjà récipiendaires de l'obligation déclarative préalable. La réception d'une déclaration préalable et l'instruction d'un régime d'autorisation sont pourtant deux choses distinctes. Si cette disposition s'appliquait, les Safer, qui sont, je le rappelle, des sociétés de droit privé, se verraient confier la réception de la déclaration et la vérification et l'instruction du dossier. Il paraît exorbitant du droit commun qu'elles instruisent « au nom et pour le compte de l'autorité administrative ». Pour des raisons d'indépendance, l'autorisation administrative doit émaner complètement de l'État et être instruite par ses services. Quel est l'avis de la commission

la procédure du dispositif de contrôle pour permettre l'instruction des dossiers par les services préfectoraux à la place des comités techniques des Safer, lesquels pourront toutefois se voir déléguer cette instruction. Si je partage sans réserve cette volonté de clarifier les rôles de chacun et de maintenir l'indépendance de l'autorité administrative, les différentes auditions que j'ai menées, y compris auprès des services préfectoraux, m'ont m'ont convaincu de la nécessité de conserver l'instruction des dossiers par les comités techniques des Safer, qui disposent des compétences pour ce faire. Dans les faits, ma chère collègue, la délégation aux Safer que vous proposez sera systématique. par ailleurs à vous rassurer, car la commission des affaires économiques a adopté plusieurs modifications du texte permettant, tout au long de la procédure, de clarifier les rôles de chacun et de mieux encadrer l'extension des prérogatives des Safer.

l'avis du Gouvernement ?

et d'orienter le foncier vers les projets les plus conformes à nos orientations politiques, professionnelles et territoriales en matière d'installation et de consolidation des exploitations. Faute d'un seuil adapté, le contrôle prévu dans la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vidé de ses effets.

Le texte issu de la commission des affaires économiques a en effet encore élargi ce champ, désormais compris entre deux et quatre fois la Saurm fixée dans le SDREA. Ce seuil semble totalement déconnecté des objectifs de lutte contre la concentration excessive et l'accaparement

Comme nous aurions aimé pouvoir le défendre en présentant notre amendement n° 73, nous souhaitons aligner le système de contrôle des sociétés sur le système actuel de contrôle des structures. Le présent amendement est donc un amendement de repli qui vise à maintenir dans la

utile régionale moyenne. L'auteur de la proposition de loi n'a pas choisi ce seuil au hasard, mais à l'issue de nombreuses consultations au sein du monde agricole. Un équilibre a été trouvé pour que le contrôle se déclenche à un niveau rendant le dispositif pertinent. Libre au préfet de décider ce qui est souhaitable, au vu de la réalité du foncier agricole et des types d'exploitation de sa région : ce qui est excessif ici, pour la pomme de terre, ne le sera pas forcément là, pour la vigne. Le défi de la transmission impose dans tous les cas un contrôle relativement serré de l'agrandissement des exploitations sous forme sociétaire.

: faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. Or la commission des affaires économiques a encore accru le seuil plafond à quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne, tout en étendant le champ des exemptions. Cette rédaction creuse encore l'inégalité de traitement que subissent les autres modes d'accès au foncier agricole, soumis, eux, à un

Il ne faudrait pas que cette proposition de loi soit pire que la situation actuelle. Nous devons préserver nos terres agricoles et les exploitations à taille humaine, mais aussi faire en sorte que nos agriculteurs soient présents sur leurs exploitations, car ce sont eux qui font vivre nos territoires et entretiennent nos savoir-faire, et non de grandes sociétés qui vivent de la spéculation et du rendement.

tout en garantissant une certaine fluidité des transactions sociétaires sur le marché foncier agricole. Or un seuil plancher inférieur à deux fois la surface agricole utile régionale moyenne permettrait de contrôler les exploitations dont la surface se situe tout juste dans la moyenne régionale, ou juste au-dessus

Il s'agit ici de déterminer quel sera le seuil retenu pour le déclenchement du contrôle quand la société se situe hors du territoire français ou lorsque le siège social n'est pas dans la même région que celle du lieu d'exploitation.

Le lieu du siège social est peu représentatif de cet impact ; de surcroît, sa modification au profit d'une zone où le seuil de déclenchement du dispositif serait susceptible d'être plus haut pourrait donner lieu à détournement.

pour les sociétés dont le siège social ne se situe pas à proximité des terres convoitées dans le cadre de la prise de contrôle. La référence au lieu où se situe la majorité des terres de la société nous semble plus adéquate à l'esprit de la procédure visée. Quel est l'avis de la commission

qui s'appliquera à l'opération. Or le texte ne précise pas, en l'état, si c'est l'implantation de la société bénéficiaire ou celle de la société cible qui est prise en compte. Cet amendement vise à acter cette précision.

Par exemple, si une société agricole basée en Normandie fait l'acquisition d'une société détenant des terres agricoles en Bretagne, il est logique que la concentration de terres qui en résulte soit appréciée au regard du seuil défini pour la Bretagne, et non pour la Normandie. Cette clarification me semble nécessaire et bien ciblée. Avis favorable.

est à M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 13, introduit en commission, qui crée une nouvelle dérogation permettant de pondérer à la hausse le seuil d'agrandissement significatif en fonction du nombre d'exploitants actifs dans la société procédant à l'opération.

Une telle modification me semble souhaitable, car elle s'inscrit dans la logique retenue par la commission : favoriser ceux qui travaillent la terre et mettent en valeur l'exploitation depuis longtemps tout en apportant les garanties nécessaires pour éviter les dérives.

Or seules les surfaces destinées à l'activité agricole doivent être comptabilisées, afin que le dispositif de contrôle soit cohérent avec les objectifs de lutte contre la concentration excessive des terres agricoles. On ne peut pas inclure

inclut notamment les surfaces classées en zone naturelle au sein d'exploitations agricoles, mais ne pouvant être cultivées, ou encore les terres protégées dans le cadre du programme Natura 2000, telles que les pelouses sèches, en raison de leur intérêt pour la biodiversité. Ces surfaces n'étant pas exploitées, il n'est pas pertinent de les caractériser comme surfaces agricoles lorsqu'on mesure l'étendue d'une exploitation agricole ou d'une société de propriété agricole. Parmi elles figurent elles figurent des surfaces agricoles qui ne procurent aucun revenu agricole ni aucune valeur économique à l'exploitation

luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. C'est pourquoi, sans supprimer totalement cette exemption, démarche qui n'aurait aucune chance d'aboutir, nous proposons de la limiter aux cessions de titres sociaux réalisées à titre gratuit en deçà du deuxième degré de parenté. Il s'agit de lutter contre tout abus ou tentative de contournement du dispositif tout en préservant une agriculture familiale. Cet amendement de repli vise à encadrer l'exemption prévue pour l'ensemble des opérations réalisées à titre gratuit. En effet, si ces opérations passent sous les radars, elles risquent fort de devenir une voie privilégiée de contournement. C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu l'auteur de la proposition de loi dans un premier temps. Comme le souligne la Confédération paysanne, la prise de contrôle d'une société peut passer par la prise de participation par acquisition de titres sociaux, mais aussi par la modification de la répartition des droits de vote. Les conventions en matière de droits de vote réalisées à titre gratuit doivent donc être soumises

un refus. Tout l'intérêt de ces dispositifs de contrôle est là : permettre d'examiner les projets présentés et leur adéquation avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires afin d'identifier de potentielles tentatives de contournement des systèmes de régulation. Merci, Cet amendement vise à revenir sur un affaiblissement de la proposition de loi voté en séance publique par l'Assemblée nationale et conforté par notre commission des affaires économiques. économiques. Sont désormais exclues du contrôle les opérations familiales réalisées à titre onéreux jusqu'au quatrième degré inclus, sous réserve du maintien de l'usage ou de la vocation agricole de l'exploitation.

au renouvellement des générations. Par exemple, on constate parfois que des exploitants agricoles ont pu bénéficier de la priorité à l'installation pour acquérir des terres et qu'ils ont, quelques années plus tard, repris une autre

: une demande d'autorisation d'exploiter n'engendre pas nécessairement un refus. Elle permet de s'assurer de l'adéquation des projets présentés avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires. En supprimant cette exemption,

les cessions de parts sociales ou d'actions entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. En effet, l'une des réponses trouvées par le monde rural l'accès à la propriété et permettre la transmission du foncier a été de capitaliser sur la diversité et la richesse des liens familiaux au sein des groupements fonciers agricoles (GFA). Nous entendons préserver cette capacité d'action dans le cercle familial élargi

un décès. Afin de préciser le champ d'application de l'exemption et de sécuriser les transmissions familiales- enjeu majeur pour la pérennité de l'activité agricole en France et le renouvellement des générations en agriculture

face aux effets potentiellement problématiques d'une concentration excessive des terres. Les termes adoptés sont donc trop vagues et nous exposent à de nombreux contentieux. Pour ces raisons, il nous paraît important de rétablir la version selon laquelle le demandeur peut bénéficier de l'exemption familiale s'il exploite personnellement les terres

installations, de la préservation des terres ou de la lutte contre les concentrations excessives.

Cet amendement vise à revenir sur de nouvelles exemptions au dispositif de contrôle prévu par le présent texte.

depuis au moins neuf ans et inscrits dans un parcours d'installation ou dans le répertoire départemental d'installation. Nous reconnaissons que cette nouvelle dérogation vise un objectif plus noble que les précédentes,

Premièrement, cette discussion commune porte sur le principe même des exemptions. Je considère qu'il est très important de maintenir la fluidité des transactions sociétaires sur le marché foncier agricole et que le dispositif prévu par cette proposition de loi n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des opérations.

Deuxièmement, cette discussion commune porte sur l'exemption des cessions réalisées à titre gratuit. Il est proposé de la restreindre aux cessions entre proches parents. À mon sens, de telles modifications porteraient atteinte de manière injustifiée aux successions et à la liberté de transmettre son patrimoine. Je suis donc défavorable aux amendements n 80 rectifié, 53 et 164, tendant à restreindre cette exemption en fonction de la proximité du lien de parenté. Troisièmement, cette discussion commune porte sur les modalités d'application de l'exemption familiale.

vous aviez été nombreux à soutenir cet élargissement, et j'estime indispensable de le maintenir pour garantir la fluidité des transactions familiales et préserver les exploitations familiales.

et non des titres sociaux acquis depuis les neuf dernières années. Cette durée étant particulièrement longue, il est proposé, notamment en cas de décès, que les bénéficiaires des parts sociétaires conservent les titres sociaux hérités jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans et qu'ils respectent les autres conditions applicables à cette exemption.

Quant à la seconde condition, nous l'avions assouplie en commission, car la notion de participation effective à l'exploitation me paraissait trop restrictive : cette condition ne serait pas remplie d'un repreneur assurant seulement la direction de l'exploitation. Ainsi, elle obligerait le repreneur à détenir le cheptel et le matériel, ou encore à habiter sur l'exploitation. En conséquence, je suis défavorable aux amendements identiques n 83 rectifié et 109, qui visent à rétablir cette condition dans sa version antérieure.

Quatrièmement, cette discussion commune porte sur les exemptions applicables aux actionnaires associés et salariés qui participent déjà à la mise en valeur de l'exploitation depuis au moins neuf ans. Mes amendements n 189 et 190 visent à apporter des clarifications rédactionnelles nécessaires à la bonne compréhension du dispositif. Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 140 rectifié, qui vise à exempter les associés ou actionnaires de la condition d'ancienneté en cas de décès, de maladie ou d'accident entraînant une invalidité totale et définitive. Ces précisions me semblent relever du bon sens. Mes chers collègues, nous sommes toutes et tous pour la défense et la pérennité de l'exploitation familiale. Les cousins germains, les conjoints

dans le contrôle des structures, l'exemption familiale existe d'ores et déjà, au troisième degré.

titre du contrôle des structures. Or vous avez adopté des exemptions familiales jusqu'au troisième degré. Pourquoi le contrôle sociétaire ne

présenter l'amendement n° 71 rectifié. Cet amendement vise à rétablir l'exemption du dispositif de contrôle pour les sociétés foncières agricoles solidaires qui accomplissent un travail clairement identifié de préservation, de lutte contre la déprise agricole et contre la concentration des exploitations.

activité d'acquisition et de gestion par bail rural ou encore rendre un service d'intérêt économique général. Nous renvoyons à ces conditions, qui servent de garde-fous.

voir retardées leurs opérations qui suivent des objectifs vertueux conformes à leur objet social.

le rapporteur, si vous aviez opté pour une limitation globale de l'ensemble des dérogations, la suppression de cet alinéa aurait pu s'entendre. Nous aurions même pu comprendre votre démarche. Mais ce n'est pas du tout le cas et- vous en conviendrez -nous ne pouvons pas vous suivre sur ce terrain. Au-delà de ces considérations politiques, il semble indispensable de défendre le fonctionnement et le développement des structures solidaires, dont l'objet social est la préservation de la terre agricole et la lutte contre la concentration foncière, en promouvant des exploitations à taille humaine et des modes d'exploitation durables, qui allient les performances économiques, sociales et environnementales tout en favorisant l'installation et la consolidation d'exploitations existantes. Cet amendement vise donc à rétablir la dérogation supprimée en commission des affaires économiques pour les sociétés foncières agricoles d'utilité sociale.

avec l'objectif de la proposition de loi, il vise à mieux réguler le marché foncier en encadrant l'action des structures sociétaires afin de mieux préserver les terres agricoles. À cette fin, l'Assemblée nationale avait voté une exemption du dispositif au profit des foncières agricoles agréées « entreprises solidaires d'utilité sociale

Nous ne comprenons pas le choix de la commission des affaires économiques en direction de cette association. Il entre en contradiction avec l'esprit qui nous animait lors de l'examen du projet Nous avions alors tous voté un amendement du rapporteur général, notre collègue Albéric de Montgolfier, en faveur d'une réduction d'impôts pour les investissements au sein des foncières solidaires chargées d'un service d'intérêt économique général.

parallèle, toutes les sociétés agissant sur le marché foncier agricole sont soumises au contrôle de l'agrandissement significatif. Deuxièmement, cette société réalise la plupart de ses acquisitions par l'intermédiaire des Safer, dont les opérations sont déjà exemptées du dispositif de contrôle. contrôle. Troisièmement, elle met à bail les terres acquises aux seuls agriculteurs actifs en exploitation biologique. Or il n'est pas opportun, dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, de favoriser un type d'agriculture plutôt qu'un autre. Notre agriculture n'a de sens que dans la richesse et la diversité de ses systèmes de production. La commission émet donc un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques. Quel est seule. Monsieur le ministre,

de ne pas mettre en avant un système de production agricole plutôt qu'un autre ? C'est ce que vous faites ! Reconnaissons qu'en France tous les systèmes de production sont vertueux.

Merci,

Merci,

qui parlait de nature cultivée, et qui a vu mourir Claude Lévi-Strauss, ce grand ethnologue qui parlait du « phalanstère rural ». La ruralité ne s'est pas construite sur une idéologie, qu'elle soit capitalistique ou solidaire.

qui permettraient de cautionner des agrandissements excessifs au motif que quelques hectares seraient laissés à un porteur de projet. De plus, ces mesures compensatoires correspondent à des engagements à tenir après la vente, ce qui semble ouvrir la voie à des contentieux et à une insécurité juridique. Autre point problématique, la sanction envisagée en cas de non-respect de ces mesures ne semble pas suffisamment dissuasive. Nous souhaitons donc supprimer cette possibilité de compensation.

de l'État, ce silence pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient mérité une plus grande vigilance. Aussi, nous proposons de simplifier la procédure et de la rendre plus équitable. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la Safer, le représentant de l'État se prononcerait sur l'autorisation ou le refus de l'opération au regard des objectifs des le silence de l'État vaudrait refus. L'équilibre entre l'autorité de l'État et l'agilité permise par la délégation de mission d'intérêt public, les Safer,

Les auteurs de cet amendement proposent une réécriture globale proche de la procédure administrative d'autorisation préalable.

la demande d'autorisation préalable doit être déposée auprès de la Safer au nom et pour le compte de l'autorité administrative, et non pas directement auprès des services préfectoraux. Dans tous les cas, les Safer se voient notifier les transactions sociétaires, ce qui permet de ne pas demander les mêmes informations deux fois.

aux motivations des décisions prévues dans le cadre du contrôle de structure. De plus, nous réitérons notre opposition à toute mesure compensatoire et à la procédure mise en place, qui ne permettra pas à l'administration d'effectuer son contrôle dans des conditions acceptables. Nous l'avons dit, les critères pour le déclenchement de la procédure d'autorisation ne permettront de contrôler que peu d'opérations. surcroît, l'on accepte les concentrations excessives contre l'engagement de prendre quelques mesures compensatoires, c'est tout l'édifice, par ailleurs complexe, prévu par le texte qui perd sa raison d'être. Pis, ce système de dérogations et de compensations revient à légitimer l'agrandissement et le phénomène sociétaire. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. La Coalition foncière, qui regroupe de nombreuses associations, mais aussi des universitaires,

Cet amendement de repli vise à supprimer le mécanisme dérogatoire de mesures compensatoires, qui permettrait à certains d'obtenir une autorisation de prise de contrôle malgré la constatation d'un phénomène d'accaparement de terres. Les mesures de compensation peuvent être mises en oeuvre après l'autorisation du projet, ce qui pose un problème de sécurité juridique. Ainsi, selon la communication interprétative de la commission sur l'acquisition de terres agricoles et le droit de l'Union européenne, les solutions autres que les régimes d'autorisation préalable risquent de ne pas offrir la même sécurité juridique aux transactions foncières. Par exemple, des mesures postérieures au transfert, comme son annulation, compromettraient la sécurité juridique, laquelle revêt une importance fondamentale dans tout régime de transfert de terres. Ainsi, la possibilité de compensation porte en elle le risque d'offrir un blanc-seing à l'accaparement, contre la promesse de libérer quelques hectares

introduit par le présent texte, précise que toute opération réalisée en violation de cet article sera nulle. Cette nullité pourrait être exercée par l'autorité administrative. Toutefois, l'action en nullité sera prescrite dans un certain délai. Les députés l'avaient fixé à douze mois, contre cinq En commission, le rapporteur a de nouveau réduit ce délai à six mois, estimant qu'il était nécessaire de « favoriser une action rapide et d'inciter l'administration à réagir en cas de manquement aux engagements ». et si l'administration n'était pas en mesure d'instruire tous les dossiers dans un délai de six mois, la réduction du délai reviendrait, au contraire, à limiter la possibilité d'invoquer cette nullité.

à préciser que ce délai de six mois court à compter de la prise de contrôle de la société. N'oublions pas que, dès l'instant où il y a vente d'une société, il y a publicité ! Tout le monde sera donc au courant que cette société a été vendue,

Il n'est pas forcément nécessaire que ces délais soient identiques. Au contraire, si l'autorité administrative constate une cession illégale après l'expiration du délai de prescription pour engager une action en nullité de l'opération, elle doit toujours pouvoir disposer de la faculté de sanctionner, y compris financièrement,

C'est pourquoi la commission des affaires économiques avait adopté un amendement tendant à indiquer que le contenu, le format et les modalités de transmission des demandes d'autorisation seront précisés par décret. Dès

Il s'agit d'un amendement de transparence et de simplification, dont l'adoption permettra de dissiper toute incompréhension des acteurs dans le cadre de la procédure d'autorisation. Ainsi, ces derniers disposeront tous de la même information. est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction des dispositions relatives aux avis des interprofessions. La rédaction adoptée en commission prévoyait une remise obligatoire de ces avis, formulation était trop restrictive : elle aurait pour effet de bloquer la procédure d'instruction, même dans les cas où l'interprofession ne souhaite pas donner un avis sur l'opération. Cet amendement tend à offrir une formulation plus souple, aux termes de laquelle la Safer est tenue d'informer les interprofessions que celles-ci peuvent lui remettre un avis sur l'opération. Elles peuvent ensuite lui transmettre des observations, ou ne pas le faire si elles estiment

par l'exigence d'une formalité supplémentaire à accomplir auprès de ces organisations en vue de recueillir leurs observations. D'autre part, il tend à sécuriser juridiquement l'instruction conduite par les Safer et le traitement par l'autorité administrative

La proposition de loi Sempastous, que nous examinons, vise à réguler l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires ; c'est à saluer, car elle répond à une carence bien réelle de la régulation du marché foncier agricole, carence qui crée un risque d'accaparement et de concentration des surfaces agricoles. en compte les spécificités territoriales et la diversité des projets qui peuvent être défendus par les acteurs locaux, l'Assemblée nationale a introduit la possibilité pour les organisations interprofessionnelles régionales concernées de transmettre un avis facultatif

aussi de créer des situations de conflit d'intérêts lors d'opérations d'acquisition de foncier le marché sociétaire. Il est donc préférable de restaurer le caractère consultatif de l'avis des interprofessions. Les deux amendements

Il faut s'assurer que la Safer et le préfet, dans leurs rôles respectifs d'instructeur et de décisionnaire, disposent de l'ensemble des informations relatives aux exploitations et aux enjeux économiques sous-jacents.

procédure, mais aussi directement au préfet si elles le souhaitent. L'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure d'autorisation disposeront ainsi de la même information.

séance maintenant. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010 prise pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable,